Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, selon les derniers chiffres de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, 88 % des victimes d'agressions sexuelles ou de viols ne portent pas plainte. en cause le sentiment de honte et le surencombrement des commissariats, l'attente interminable au poste de police, la mauvaise formation des agents au recueil de la parole des victimes et le mauvais accompagnement qui s'ensuit. Si des formations spéciales

Des centaines de témoignages ont aussi été collectés sur le site « payetapolice.tumblr.com », afin de dépeindre le climat délétère qui règne au sein des commissariats. Aujourd'hui encore, on s'étonne et on reproche aux victimes de ne pas porter plainte ou de sortir du silence bien trop tard.

déposition. C'est une première réponse positive adressée aux victimes, accompagnées ou non par un proche ou un professionnel : elles peuvent, depuis leur domicile, prendre leur temps et passer le cap, parfois douloureux, du dépôt de plainte. Toutefois, si la dématérialisation

les personnes peuvent être accompagnées « chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure », donc pas seulement quand elles se constituent parties civiles.

demander, dès ce stade, à être accompagnées d'un avocat.

et qui n'est pas informée des finesses de la procédure se voit souvent proposer de faire une déclaration

que les victimes soient informées à chaque stade de la procédure de la situation du mis en cause, en particulier lorsque celui-ci est remis en liberté sous contrôle judiciaire ou lorsqu'il sort de détention. En effet, les victimes ne sont pas systématiquement

Vous demandez que la victime de violences conjugales soit informée à toutes les étapes de la procédure pénale. Or c'est écrit explicitement dans l'article 10-2 du code de procédure pénale.

mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions [de] l'article 138. Cette dernière en est avisée

Théophile. Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour les agents de police judiciaire adjoints(APJA), de constater le nouveau délit d'outrage sexiste aggravé. Cette possibilité, introduite par la commission des lois, des lois, présente une fragilité constitutionnelle. En effet, dans sa décision du 20 mai 2021 relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, les juges de la rue de Montpensier ont déclaré contraire à l'article 66 de la Constitution la possibilité de constater des délits pour les agents de police municipale et les gardes champêtres, qui sont des agents de police judiciaire adjoints au sens de l'article 21 du code de procédure pénale. Afin d'éviter tout nouveau risque de censure par le Conseil constitutionnel, je vous invite, mes chers

Si nous ne voulons pas que la réforme prévue à l'article 7, qui vise à renforcer la répression d'outrage sexiste, ne soit pas contre-productive, il nous paraît important que les personnes constatant aujourd'hui l'outrage sexiste puissent continuer de le faire, même si l'outrage sexiste aggravé devient un délit.

Il nous semble que pour ce « petit »- pardon du qualificatif -délit d'outrage sexiste aggravé, puni d'une simple amende, il n'est pas excessif de leur reconnaître cette compétence.

Monsieur le ministre,

de cette condition cumulative. Il peut arriver que des violences n'aient pas encore été commises ou, du moins, que la victime ne puisse pas en apporter la preuve,

monsieur le ministre,

de vos convictions sur ce sujet. Siégeant moi-même à la délégation aux droits des femmes depuis maintenant quelques années, auprès, notamment, de la présidente Annick Billon, je sais l'importance que vous accordez à ces sujets et je crois faire partie de ceux qui y sont particulièrement attentifs. Le Sénat et la commission des lois nomment des rapporteurs sur un texte

les deux rapporteurs n'ont pas mené les auditions nécessaires. Je rappelle, et je prends à témoin Jérôme Durain, que les auditions sont ouvertes aux membres de la commission des lois et que de nombreux collègues y ont participé. Nous sommes obligés de maintenir une certaine méthode dans l'examen de ce texte.

d'après les chiffres publiés par votre ministère en janvier dernier, les violences physiques contre les édiles ont augmenté de 47 % sur les onze premiers mois de 2021, par rapport à la même période de l'année précédente. Derrière ces statistiques, ce sont exactement 1 186 élus qui ont été pris pour cibles et 419 outrages qui ont été recensés. Or seule une poignée d'agressions verbales et physiques envers les élus de la République connaissent des suites judiciaires et quand bien même une procédure judiciaire est enclenchée, l'on n'enregistre en réalité qu'un très faible nombre de condamnations, même en cas d'agression physique. La plupart du temps, les plaintes sont classées sans suite ou ne font l'objet d'aucune suite pénale.

On l'a bien compris : l'article 7 vise à réprimer plus sévèrement les refus d'obtempérer, en alourdissant la peine encourue et en diminuant les crédits de réduction de peine auxquels peuvent prétendre, pour bonne conduite, les personnes condamnées à une peine privative de liberté après avoir commis cette infraction.

je pense que Mme Delattre a tout à fait raison. De plus, selon les remontées de l'ensemble des centres de veille du ministère de l'intérieur, 1 037 procédures établies impliquant un élu comme victime ont été constatées, dont 157 pour violence physique et 808 pour menace ou outrage.

Notre groupe va prendre ses responsabilités. Nous sommes extrêmement attachés à la défense de l'exercice du mandat d'élu, mis en cause

Premiers représentants de l'État dans nos communes, ils doivent être mieux protégés dans leurs fonctions. En réponse à l'escalade du nombre d'agressions, il appartient à la représentation nationale de contribuer à ce que leur figure d'autorité soit pleinement réintégrée dans l'esprit collectif. Les plaintes qu'ils peuvent déposer dans ces circonstances font régulièrement l'objet de classements sans suite, qui, sans préjuger de leurs motifs profonds, conduisent à renforcer de leurs motifs profonds, conduisent à renforcer le sentiment d'abandon des maires et des élus locaux face aux violences dont ces derniers peuvent être victimes. Cet amendement vise donc à rendre systématique la procédure de composition pénale, procédure de substitution à la poursuite prévoyant le versement d'une amende, préalablement à tout classement sans suite, dans le cadre d'une procédure d'agression physique ou verbale d'un élu dans l'exercice de son mandat. Ainsi, aucune plainte d'élu en la matière ne resterait sans réponse.

telle solution est donc limitée aux cas pour lesquels le classement sans suite pourrait être envisagé. La circulaire du garde des sceaux de septembre 2020 a marqué une étape vers une meilleure réponse pénale ; nous y contribuons aussi, dans le cadre de ce texte, en renforçant les sanctions.

de leurs fonctions, ou en raison de celles-ci, mais concernent également les membres de leurs familles. Fort de ce constat, Éric Gold avait déposé en octobre 2019 une proposition de loi visant à lutter contre les incivilités, menaces et violences envers les personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public, afin de renforcer la réponse pénale en cas d'agressions d'élus ou de dépositaires de l'autorité publique. Cet amendement reprend l'article 1 de cette

Les marches blanches organisées par les familles et la population en hommage aux victimes de violences gratuites s'enchaînent, les slogans « plus jamais ça ! » se succèdent, en vain Redoine, Adrien, Grégory, Sofiane, Kevin, Thomas ont été défigurés pour un refus de cigarette, poignardés pour avoir doublé une voiture dans une station d'essence, frappés à mort pour une place de parking ... Ces actes commis sur la voie publique

se sont trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Lors du discours de politique générale qu'il a prononcé à l'Assemblée nationale le 12 juin 2019, le Premier ministre Édouard Philippe avait réaffirmé la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre un plan pour lutter contre ces violences gratuites. « Nous ne devons plus rien

En première analyse, on ne peut que s'interroger sur les conséquences que l'adoption d'un tel amendement emporterait sur la tenue du procès pénal : ne risque-t-on pas d'assister à des discussions byzantines pour savoir si la réaction de l'auteur des faits était proportionnée ou pas ? Le procès ne risque-t-il pas de dériver vers une analyse du comportement de la victime, pour apprécier si celui-ci constituait ou non une provocation ? Ces questions justifieraient que nous entendions des universitaires

monsieur le ministre,

l'approche statistique qui nous est présentée. Les policiers et les gendarmes tirent plus que dans d'autres pays et ils tirent plus sur des véhicules.

commission ? Les conditions d'usage des armes en cas de refus d'obtempérer ont été précisées par le législateur au début de l'année 2017, après un dialogue nourri entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui a abouti à une formulation équilibrée tenant compte des exigences du maintien de l'ordre, tout en limitant le recours aux armes à feu au strict nécessaire. Le code de la sécurité intérieure prévoit que l'usage des armes est autorisé lorsque policiers et gendarmes « ne peuvent immobiliser autrement [ ...] des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ». Cet amendement tend à effacer le compromis trouvé à l'époque, pour revenir à la rédaction initiale du projet de loi déposé par le Gouvernement, plus restrictive encore pour les forces de l'ordre. Ce n'est pas la direction dans laquelle nous souhaitons nous engager ; l'avis de la commission est défavorable.

Merci